de l'article. Sous couvert de simplification et de nouveauté, le présent texte apporte parfois des modifications dont on peine à comprendre la justification et le réel intérêt. C'est le cas de cet article 6,

Cela n'empêche nullement le Gouvernement, en cas de nécessité, de proposer des mesures fiscales dans un texte ordinaire, comme il l'a fait en décembre 2018, voire de présenter une loi de finances rectificative. C'est donc surtout un signal utile. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Ainsi

fait de la loi de fin de gestion une loi d'ajustement. Cela n'empêchera jamais un gouvernement de déposer une véritable loi de finances rectificative, comprenant éventuellement des mesures fiscales. Quoi qu'il en soit, pour nous, la loi de fin de gestion est vraiment un exercice d'ajustement. Nous sommes donc très favorables à la rédaction du texte en l'état, et par conséquent défavorables à l'amendement du sénateur Delahaye. Monsieur Delahaye, l'amendement

tout en préservant la qualité et l'exhaustivité de leur contenu. En l'état du droit, la transmission est prévue cinq jours francs avant l'examen des crédits concernés. Le texte de la proposition de loi organique vise à avancer cette date au premier mardi d'octobre.

des instituts français de recherche, qui sont placés auprès de nos postes diplomatiques et consulaires, s'appuie sur un statut d'établissements à autonomie financière, ou EAF, créé par la loi de finances de 1974.

ces établissements à autonomie financière devaient être supprimés, nous perdrions une énorme capacité de flexibilité pour le fonctionnement de nos instituts français à l'étranger, qui, aujourd'hui, grâce

sans que l'avenir de nos établissements à autonomie financière à l'étranger soit remis en cause. Nous vous proposons donc un dispositif permettant de prendre en compte les spécificités et les besoins de nos établissements à autonomie financière, en particulier de nos instituts français, en les inscrivant clairement dans la LOLF, tout en prévoyant un moyen et un dispositif d'information du Parlement sur l'ensemble de l'activité de recette des instituts français à l'étranger. S'il apparaissait que ce dispositif doit encore être amélioré techniquement, nous pourrions nous en remettre à la seconde lecture

monsieur le ministre,

cela fait maintenant des années que tout le monde bute sur ce sujet, avec la volonté de protéger et de garantir le statut des élèves. C'est la raison pour laquelle, sans préjuger

la volonté d'inscrire une obligation annuelle pour le Parlement de débattre sur la dette de fait, une orientation politique. Certes, la dette est un sujet important, dont nous débattons régulièrement à chaque projet de loi de finances. Nous en avons discuté l'année dernière au cours d'un débat organisé sur l'initiative du groupe Les Républicains. La commission des finances a mené des auditions et a organisé des tables rondes. Le débat a été intense dans le monde économique et dans le domaine de la recherche.

Il s'agit d'être cohérent dans le temps. Nous essayons au Sénat de l'être, à défaut que d'autres le soient- je fais référence à mon intervention de tout à l'heure, monsieur le ministre, car je n'en démords pas

et aux souscripteurs au cours d'une année des titres émis, on a du mal à obtenir des informations précises, y compris le rapporteur spécial, qui vient de s'exprimer sur le sujet.

traite à la fois les perspectives d'évolution du financement de la dette et les prévisions de recettes des administrations publiques. Les débats et le vote du Parlement ne sauraient se centrer sur les seules dépenses. Ils doivent incorporer une prise en compte éclairée des perspectives de recettes existantes. Tel est l'objet de cet amendement.

Un certain nombre de banques centrales nous ont fait savoir qu'elles n'appréciaient pas que nous fournissions autant de détails. Elles n'avaient pas envie que tous leurs investissements soient rendus publics de la sorte

Si la banque agit pour le compte d'un établissement situé dans l'Ohio, qui travaille lui-même pour le compte de quelqu'un situé dans les îles Caïman ou dans le Delaware, il sera très compliqué de s'assurer du respect des règles standard et de ne pas se trouver dans un paradis fiscal. En l'état actuel, je ne puis vous dire si c'est le cas ou non. » Au nom de la dette, on nous impose depuis des décennies la réduction des dépenses publiques la compression des dépenses utiles à la société. La transparence est un minimum, et une action reste à mener pour savoir qui détient notre dette

la dette publique, pour une part non négligeable, fait l'objet d'un marché secondaire, sur lequel un titre peut changer de détenteur plusieurs fois

l'acquisition de la dette sur tel ou tel créancier, dans la mesure où, de manière générale, lorsque nous émettons des obligations, le taux de couverture

J'ajoute que la publication de la totalité des possesseurs de la dette serait extrêmement difficile, à la fois pour les raisons évoquées par M. le rapporteur, qui concernent la multiplication des opérations et leur rythme infra-annuel, et parce que des particuliers se retrouvent investisseurs dans la dette française : nous estimons à 2 millions le nombre de particuliers qui, directement ou indirectement, auraient des titres ayant trait à la dette française, ce qui rendrait la publication tout à fait impossible techniquement.

Une autre étude récente montre que la France épuise l'intégralité de son budget carbone annuel entre les mois de janvier et de mars. Le reste de l'année civile, nous vivons à crédit sur le climat.

argument que l'on peut entendre, même si j'ai dit précédemment que nous n'avions pas prévu de trajectoire pour les recettes. Or, pour corriger l'absence de compteur des écarts sur les recettes, vous nous proposez de supprimer le compteur d'écart sur les dépenses !

est à M. le rapporteur. Cet amendement tend à faciliter l'exploitation des informations figurant dans les annexes au projet de loi de finances, tout particulièrement dans les projets annuels de performance. Nous nous inspirons d'une disposition similaire introduite par la commission des affaires sociales, sur la proposition de son rapporteur, dans la proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Il s'agit d'un accès sous forme de fichier informatique aux données contenues dans les documents annexés au projet de loi de finances. Quel est l'avis du Gouvernement ? projet de loi de finances. Quel est l'avis du Gouvernement ? D'un point de vue juridique, cette mesure ne relève pas du législateur organique, dans la mesure où il s'agit simplement d'un format de données. Pour autant, je précise que la transmission des données demandées ne pose pas de difficultés sur le fond et que le Gouvernement peut s'engager à ce que les données présentées dans les annexes au projet de loi de finances soient transmises au Parlement dans un format exploitable, dans la limite des formats disponibles sur les applications interministérielles utilisées par les administrations. J'indique, pour être tout à fait complet, que je ne peux pas m'engager aussi largement pour la totalité du PLF pour 2022, du fait de l'état d'avancement des travaux. En revanche, je m'engage, au nom du Gouvernement, à ce que l'intégralité des données pour le PLF pour 2023 soit transmise et à ce qu'un maximum de données pour le PLF pour 2022 le soit aussi. Au regard de cet engagement, je sollicite donc le retrait de cet amendement.

fiscalité. Cet amendement vise à prévoir un débat sur la base d'un rapport qui prendrait en compte l'ensemble des sources de financement de l'intervention publique. Quel l'avis de la commission ? Le tableau d'équilibre présente le montant des dépenses, ainsi que l'estimation des produits des ressources fiscales et des ressources non fiscales. Le financement de la dépense, plus précisément du solde entre les dépenses et les recettes, est précisé par le tableau de financement qui figure dans le même article. Il semble donc que tous les éléments sur lesquels porte la demande de publication d'un rapport dans cet amendement

Mais cela n'est pas possible, puisque les recettes sont versées au budget général, sans être affectées à des dépenses particulières, sauf dans le cas limité des taxes affectées. C'est la raison pour laquelle je demande le retrait

Mme Isabelle Briquet. Le coût des dépenses fiscales en France représente environ 100 milliards d'euros annuels. Si les niches fiscales ne doivent pas être combattues par principe, elles doivent être mieux encadrées et contrôlées par le Parlement. Dans cette perspective, il n'est pas acceptable que, comme l'a rappelé la Cour des comptes en 2019, un tiers des dépenses fiscales aujourd'hui ne soit pas évalué. L'objet du présent amendement est donc de créer un dispositif qui permette de renforcer l'évaluation des dépenses fiscales, sans pour autant nier leur utilité. En pratique, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne fournirait pas au Parlement durant quatre années consécutives une évaluation, les dépenses les dépenses fiscales en question seraient automatiquement et obligatoirement abrogées. Il appartiendra donc à l'exécutif de faire en sorte que les dépenses fiscales qui ont apporté la preuve de leur efficacité puissent perdurer. Conscients du travail important que représente un tel changement de paradigme, les auteurs du présent amendement proposent une application au 1 janvier 2025, afin de laisser au Gouvernement suffisamment de temps pour mettre en place les dispositifs adéquats. Quel est l'avis de la commission ?

ce qui permet de vérifier que les objectifs fixés sont atteints et que ces dépenses restent pertinentes, tout en en mesurant le coût. Néanmoins, une suppression automatique après quatre ans me semble porteuse de risques et d'insécurité juridique,

D'une certaine manière, c'est ce que nous faisons, même si ce n'est pas ici un compteur des écarts. Nous disons qu'il faut aussi parler des recettes. Les niches fiscales représentent 100 milliards d'euros par an.

évaluation de son efficacité. Puis, au mois de juin dernier, est sorti un rapport de France Stratégie remettant en cause l'efficacité du crédit d'impôt recherche, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Je ne

Elles sont censées être incitatives et aider à atteindre des objectifs communs. Or on a le sentiment que, bien souvent, elles ne sont pas, ou plus au fur et à mesure de leur inscription, utilisées comme des dépenses visant un certain nombre d'objectifs,

d'effectuer un contrôle de l'action gouvernementale en matière d'exécution budgétaire, rôle jusque-là exclusivement dévolu aux présidents, aux rapporteurs généraux et spéciaux de ces commissions. Le rôle de contrôle et d'évaluation de l'action publique des parlementaires est consacré dans la Constitution. La rédaction de l'article 57 de la LOLF y contrevient, et cela de la plus explicite des manières. Cet amendement tend à y remédier, pour assurer la cohérence de notre droit, afin de permettre une appréciation de l'action de l'État aussi fine que possible et pour restaurer les pouvoirs du Parlement. Choisir d'exclure des procédures de contrôle la majorité des membres de la commission des finances nous prive d'une capacité de travail impressionnante, tout en faisant fi des sensibilités de chacun et des possibilités de tous, en confiant à nos collègues, dont le temps est largement restreint au vu de leurs attributions, le soin de nous informer tous et toutes. Pour d'aucuns, la LOLF est une forme de Constitution. Nous nous élevons contre ce texte qui, non content de saper notre initiative, nous empêche aussi dans notre capacité de contrôle. Restaurer Restaurer le Parlement, c'est avant tout en respecter les membres, leur garantir une égalité minimale dans leurs attributions ; les investigations et auditions librement décidées en font partie. Cet amendement ne coûte rien- ce n'est pas un petit argument ! -, puisque nous souhaitons simplement laisser le choix à chaque membre de la commission d'effectuer des contrôles. Nous avons beaucoup discuté des marges de manoeuvre s'agissant de nos votes sur les lois de finances et de la quantité d'informations on nous abreuve à n'en plus finir. Nous souhaitons pouvoir chercher là où est l'information dont nous estimons avoir besoin pour effectuer notre mandat comme il se doit.

L'amendement que vous proposez tend à supprimer cette distinction, de sorte que chacun des membres de la commission des finances pourrait exercer ces pouvoirs pour toute question relative aux finances publiques. Cela signifierait que les ministères devraient répondre à chacun des membres de la commission sur les mêmes sujets. Cette Cette extension paraît préjudiciable à la qualité du contrôle parlementaire. La spécialisation des rapporteurs leur permet en effet d'acquérir une véritable expertise, indispensable à l'efficacité de leur travail.

rapporteur. Cet amendement vise à poser le principe d'un accès aux données de l'administration fiscale pour l'accomplissement des missions de législation, de contrôle et d'évaluation de la commission des finances. Cet accès porterait sur des données auxquelles les chercheurs ont d'ores et déjà accès, et aurait lieu notamment dans le respect des principes d'anonymisation des données. Un tel accès est en effet indispensable pour que le Parlement puisse se doter d'une capacité de modélisation et de chiffrage des propositions formulées dans le cadre des lois de finances.

Au surplus, la procédure à laquelle l'amendement vise à renvoyer a seulement vocation à s'appliquer à l'accès des tiers à des fins de recherches scientifiques aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, des droits, des taxes et des redevances prévus au code La dérogation ne peut être autorisée que par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique tenant compte notamment des enjeux attachés à la protection de la vie privée, du secret des affaires et au respect du secret professionnel, du secret fiscal, ainsi que la disponibilité des données demandées. Pour toutes ces raisons, l'avis du Gouvernement

L'amendement vise à prévoir la publication, en annexe de chaque projet de loi de finances, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées dans le texte de loi. Le code source est une traduction en langage informatique des dispositions votées par le législateur, ainsi que des dispositions réglementaires et de la doctrine qui les précisent. Dans le cadre plus spécifique de l'examen des lois de finances, cette réforme permettrait, d'une part, de clarifier l'intention du Gouvernement, dans la mesure où les dispositions législatives proposées en vigueur comportent parfois des ambiguïtés, voire des contradictions, et que leur portée effective dépend largement de mesures d'application qui ne relèvent pas du Parlement ; et, d'autre part, de tester plus facilement les réformes proposées, de retenir des hypothèses différentes et de formuler des propositions alternatives de manière rigoureuse sans forcément interroger de manière récurrente les services de Bercy, qui nous répondent dans des délais plus ou moins longs et à qui nous sommes obligés de suggérer régulièrement des modifications tout au long du processus d'élaboration de la loi. La commission des finances du Sénat avait, par exemple, mis en ligne un simulateur de la mesure proposée dans un rapport de 2017 sur la fiscalité de l'économie collaborative. La réforme proposée sera donc absolument utile au Parlement, mais aussi aux citoyens ou encore aux chercheurs. Elle nourrirait le débat public, avant et après le vote de la loi, dans une démarche d'évaluation des politiques publiques cohérente avec la réforme de la procédure d'examen des lois de finances actuellement envisagée par le Gouvernement. Cet amendement vise donc à tirer les conséquences, pour ce qui concerne le processus législatif, du principe général d'ouverture des données publiques posé par l'article 1de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. L'article 2 de cette loi a ajouté les codes sources à la liste des documents administratifs dont la liberté d'accès est garantie par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il serait donc paradoxal que les parlementaires de simulations disposer de ce que les citoyens peuvent obtenir. Les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer ces documents à toute personne qui en fait la demande. L'article 4 a quant à lui créé un principe de communication des algorithmes lorsque ceux-ci ont participé au fondement d'une décision individuelle, ce qui s'applique naturellement aux impôts. impôts. Les éléments publiés correspondraient aux documents administratifs que l'administration est d'ores et déjà tenue de publier ou de communiquer aux personnes qui en font la demande, et ne couvrent aucun document portant atteinte, entre autres, au secret des délibérations du Gouvernement ou du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la vie privée, au secret médical ou encore au secret commercial. Ils seraient publiés dans le respect de la loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Quel est l'avis de la commission ?

que l'algorithme est construit en fonction des dispositions votées par le Parlement. Dès lors que cet algorithme traduit des décisions votées par le Parlement, il est difficile d'introduire dans le rapport de présentation du PLF un algorithme qui s'appuierait sur des dispositions qui n'ont pas été encore votées et sont susceptibles d'évoluer.

Calquée sur le droit de tirage des groupes concernant les commissions d'enquête, cette mesure permettra de renforcer l'assistance de la Cour des comptes au Parlement. Cette proposition se place dans la suite logique d'autres. Les parlementaires ont toute latitude pour choisir les informations dont ils estiment avoir besoin pour contrôler l'action du Gouvernement. La production d'un rapport sur une thématique choisie se situe dans la droite ligne des attributions de la Cour, de son périmètre d'action et de ses compétences. Ce dispositif s'inscrit dans un schéma vertueux, entre le Parlement, cette institution financière et les citoyens.

Les parlementaires, en tant qu'élus du peuple ou de leurs représentants, peuvent s'intéresser à des sujets dont la Cour ne serait pas saisie. L'adoption de cet amendement aurait la vertu supplémentaire d'assurer une information constante à la Cour.

demande de droit de tirage d'un rapport auprès de la Cour des comptes, pour chaque groupe, une fois par session parlementaire. Quel ? Cet amendement a pour objet que la Cour des comptes, dans le cadre de la mission d'assistance au Parlement qui lui est confiée par l'article 47-2 de la Constitution, soit amenée à remettre chaque session un rapport sur un thème prévu par chaque groupe parlementaire.

ne porteraient pas nécessairement sur les missions attribuées à la Cour des comptes par la Constitution. Elle pourrait également conduire à la réalisation de travaux multiples sur des sujets similaires. Enfin, les rapporteurs spéciaux des commissions des finances, qui appartiennent à tous les groupes parlementaires, peuvent déjà proposer chaque

à M. le ministre délégué. L'amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de nouveaux tableaux pour récapituler, par ministère, le nombre d'emplois rémunérés par l'État. En effet, cette annexe semble redondante avec les outils de suivi des emplois existants. Dans sa rédaction actuelle, la LOLF prévoit déjà, pour chaque ministère, que soient joints au PLF des tableaux qui retracent par catégorie, par corps, par métier ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'État et la justification des variations,

Nous proposons que le mandat du Haut Conseil des finances publiques s'élargisse pour apprécier la cohérence du budget de l'État au regard du bien-être social et environnemental.

Pour autant, il ne paraît pas pertinent de confier au Haut Conseil des finances publiques la mission proposée. Le Haut Conseil a été créé afin d'offrir, dans le cadre des engagements européens,

Je cite : « Permettez-moi d'ailleurs ici de contester avec la plus grande vigueur le bien-fondé de la mise en place du Haut Conseil des finances publiques, aréopage de prétendus sages, cousin d'un Conseil constitutionnel dévolu au domaine budgétaire, dont on ne sait pas trop s'il va servir d'arbitre entre les écoles de pensée économique, pour résoudre le problème de l'effort et du solde structurels, de conseil en gestion, pour le compte de l'État, de gardien du temple de l'orthodoxie budgétaire européenne, pour le compte de la Commission de Bruxelles, ou de prescripteur d'injonctions à agir, pour un gouvernement qui se laisserait aller à mener une politique budgétaire différente. Les échanges de vues récents en commission des finances entre le président, le rapporteur général et M. Moscovici m'ont rappelé le prononcé de ce discours. Le premier président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil des finances publiques se sent légitime pour contredire les parlementaires sur leurs appréciations politiques,

ou non, de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire une importance toute particulière lorsqu'il s'agit, pour la France, de ne pas respecter les critères de Maastricht prévus par ledit article 3 ce à quoi elle s'est malheureusement habituée. Le présent amendement vise à rendre systématique la constatation par le Haut Conseil des finances publiques de l'existence ou non de circonstances exceptionnelles, afin de rendre plus sincère le débat public en la matière.

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour le Haut Conseil des finances publiques d'émettre un avis sur l'exécution de l'année en cours, lorsqu'il est saisi à l'occasion du projet de loi de finances. D'une part, le suivi de l'exécution n'est pas l'objet de la saisine sur le PLF. Le Haut Conseil des finances publiques est amené à se prononcer plus avant sur l'exécution dans le cadre des projets de lois de finances rectificatives. D'autre part, l'enjeu est ici davantage de renforcer le rôle de vigie à long terme du Haut Conseil des finances publiques que de lui donner un rôle de comité de suivi de l'exécution des recettes et des dépenses de l'année en cours. Enfin, la conformité de l'exécution budgétaire à l'autorisation parlementaire doit être évaluée par le Haut Conseil une fois l'exercice clos, et non en cours d'exercice.

de tous les documents transmis par le Gouvernement au Haut Conseil des finances publiques en vue de l'élaboration d'un avis, sur la demande des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances du Parlement.

insérées dans la LOLF sont réunies. Le Haut Conseil des finances publiques demeure libre de déclarer que tel n'est pas le cas, ce qui constitue une garantie suffisante pour éviter le risque d'un abus d'usage de cette clause de sauvegarde.

qui tendent à confier au Haut Conseil la mission de se prononcer sur la prévision d'exécution pour l'année en cours à l'occasion du projet de loi de règlement et du PLF, et de préciser par ailleurs les risques qu'il identifie. L'amendement vise

à l'amendement n° 61 de M. Rambaud. Nous considérons que les dispositions de la PPLO visent à constater les écarts par rapport à une trajectoire à la fin de l'exercice et qu'il n'y a pas lieu de doter le Haut Conseil des finances publiques d'un rôle de comité de suivi tout au long d'un exercice. Nous sommes donc très favorables à cet amendement.

sur le plan fiscal la répartition non de la charge fiscale, mais des contributions entre les différentes catégories de contribuables, pour appréhender l'équité fiscale dans la mise en oeuvre des politiques publiques.

champ encore assez neuf, mais qui relève, me semble-t-il, d'une mission essentielle pour la Haute Assemblée. La proposition qui vous est soumise s'inscrit aussi, et surtout, dans un contexte très spécifique pour les finances publiques en général et pour les finances sociales en particulier.

Ce déficit, n'en ayons pas honte ; il est le symptôme de l'effort inouï entrepris par la sécurité sociale pour nous protéger tous, lors de la crise majeure que nous avons traversée, notre système de santé, mais aussi grâce au filet de sécurité qu'elle représente.

complètement les effets durables de la baisse d'activité en 2020. Certes, la sécurité sociale est une gigantesque machine assurantielle, mais celle-ci n'est pas composée de lignes comptables abstraites ; elle est intimement liée à la vie des Français et aux épreuves que ceux-ci traversent.

pour faire face à cette situation, il faut concevoir une réponse qui s'inscrive dans la durée, et une réforme d'ampleur des lois de financement de la sécurité sociale en constitue le fondement, lequel nous permettra de reconstruire une sécurité sociale mieux assise, plus solide et plus efficace.

parce qu'il permettra, pour la première fois, de disposer en loi de financement de la sécurité sociale d'une information directement lisible et utilisable sur le solde des administrations de sécurité sociale, lesquelles recouvrent un périmètre légèrement

Cela ne doit évidemment pas nous amener à abandonner le pilotage de la sécurité sociale par les soldes, qui reste notre boussole ; toutefois, dans un contexte dans lequel les recettes ont durablement chuté et dans lequel le redressement de nos finances publiques de nos finances publiques ne doit pas passer par une augmentation des prélèvements obligatoires, les dépenses devront, de toute évidence, faire l'objet d'une attention particulière. La référence aux lois de programmation des finances publiques, qui seront adoptées au début de chaque mandat, permettra également de fixer un cap contraignant.

au printemps, la constatation des comptes échus et, surtout, un débat autour de l'évaluation des politiques financées et des résultats obtenus, et, à l'automne, l'actualisation de la trajectoire de l'année en cours et le vote de la trajectoire de l'année à venir. L'article 24 de la Constitution trouvera sa pleine effectivité dans ce nouveau calendrier, avec, à l'automne, le vote de la loi, et, au printemps, le contrôle de l'action du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques.

de texte constituent en effet les deux jambes de nos finances publiques, et l'alignement des calendriers permettra un mouvement encore plus synchrone, avec notamment une présentation conjointe des deux textes en conseil des ministres, afin de disposer d'une vision panoptique de nos finances publiques.

à la clarification des règles d'inscription de mesures ayant un impact sur les finances sociales ou aux règles de compétences en matière d'exonération de cotisations sociales. En mobilisant l'ensemble de ces instruments, les deux textes que vous examinez aujourd'hui permettront de rédiger des lois de financement de la sécurité sociale plus lisibles, ainsi que des débats mieux organisés et plus efficaces. Ils jettent ainsi les fondements d'une reconstruction de nos finances sociales, et nous pouvons collectivement nous en féliciter. Je sais que ce sont des objectifs auxquels vous adhérez largement et qui convergent avec ceux d'une proposition de loi organique déposée devant la Haute Assemblée par votre rapporteur.

dont nous discuterons, sur le texte de la commission, mais, comme vous le savez, nous sommes opposés à une extension pure et simple du champ des lois de financement de la sécurité sociale à l'assurance chômage. En effet, en l'état, cela nous semble remettre trop en question l'autonomie des partenaires sociaux en la matière. L'intégration dans le solde des administrations de sécurité sociale nous paraît constituer, à cet égard, un point d'équilibre plus satisfaisant. De même, si la règle d'or est évidemment une piste intéressante pour renforcer le pilotage des comptes de la sécurité sociale, les conditions économiques ne nous semblent pas réunies pour envisager raisonnablement l'introduction d'une telle règle dès maintenant. Certaines dispositions, plus techniques,

et le cadre d'examen des lois de financement de la sécurité sociale. Ces occasions sont rares, puisqu'il s'agit simplement de la deuxième évolution depuis la création de ces lois, voilà Le Sénat et, au premier chef, sa commission des affaires sociales l'abordent donc naturellement dans un esprit constructif. Cela fait d'ailleurs longtemps que nous avons mené, avec d'autres instances, une réflexion sur les lois

Sur ce fondement, nous avons accueilli avec bienveillance la principale mesure du texte de Thomas Mesnier, c'est-à-dire la création des lois d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Lacss), qui

Là aussi, notre proposition de loi prévoyait un tel article. Nous avons également fait bon accueil au réaménagement des annexes, dû à la création de la Lacss, ainsi qu'à la création d'annexes dédiées à la situation financière de l'assurance chômage, des régimes complémentaires de retraite et des établissements publics de santé. Là encore, nul ne devrait avoir peur de l'amélioration de l'information du Parlement en matière de finances sociales. Enfin, nous n'avons pas d'opposition à l'égard de l'évolution du calendrier, qui améliorera les conditions d'examen du PLFSS par l'Assemblée nationale. Je vous demanderai néanmoins à ce sujet, madame la ministre, deux confirmations

et, d'autre part, que le calendrier d'examen par le Sénat demeurera inchangé, avec un passage en séance aux environs de la mi-novembre Cela dit, vous le savez, madame la ministre, notre proposition de loi organique était plus ambitieuse que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, en particulier pour ce qui concerne les droits du Parlement. C'est donc, très logiquement, cette ambition que les amendements adoptés par la commission des affaires sociales ont introduite dans la proposition de Thomas Mesnier. ambition touche d'abord au périmètre des lois de financement, avec une extension à l'assurance chômage ; nous sommes là en désaccord. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point plus longuement lors de l'examen des amendements. Je tiens simplement à rappeler qu'il ne s'agit nullement de s'attaquer au paritarisme, auquel chacun connaît mon attachement personnel. Nous avons parfaitement entendu la volonté des partenaires sociaux de garder cette gestion paritaire, intégrale ou partielle, mais, il faut l'avouer, le face-à-face actuel avec le Gouvernement est déséquilibré et donne à celui-ci un pouvoir prééminent ; je comprends donc parfaitement, madame la ministre, que vous cherchiez à le conserver Nous constatons en outre que quelque 40 % du financement du régime sont issus d'une recette fiscale, ce qui me paraît naturellement impliquer le contrôle du Parlement. Nous sommes donc à la disposition des partenaires sociaux pour examiner un nouveau plan de financement de l'assurance chômage

ambition concerne ensuite le rôle normatif du Parlement en matière de finances sociales. Nous le savons tous, la LFSS n'est pas la loi de finances elle ne doit pas le devenir, et la commission des affaires sociales a d'ailleurs toujours regardé avec méfiance les idées de fusion entre ces deux textes. pour qu'un texte financier reste légitime à long terme aux yeux des Français contribuables et cotisants, il ne doit pas permettre tous les abus. les abus. Aussi, aujourd'hui comme demain, les objectifs de dépenses que nous adoptons ne doivent en aucun cas empêcher le versement d'une prestation ou le remboursement de soins à un assuré ou à un allocataire. C'est l'une des profondes différences entre les lois de finances et les LFSS, et elle doit demeurer ; nous y sommes tous très attachés. C'est la raison d'être de l'expression « objectifs de dépenses » qui figure dans la Constitution, ce que les débats au Sénat sur le projet de loi constitutionnelle de 1996 ont bien montré. En revanche, le constituant de 1996 n'a pas voulu que la sécurité sociale puisse devenir la caisse de débudgétisation du Gouvernement.

J'insiste particulièrement là-dessus, car, si les LFSS deviennent le canal commode de toutes les facilités budgétaires, elles se condamnent à terme. C'est pourquoi, sans instaurer de crédits limitatifs- j'y insiste -, nous avons renforcé les procédures de dépassement de certaines dépenses en cours d'année,

L'ambition sous-tendant nos amendements concerne également le rôle de contrôle des commissions. J'indique simplement à cet égard que, le diable se nichant parfois dans les détails, nous avons prévu que l'ensemble des données figurant figurant dans les annexes ou dans les réponses transmises par le Gouvernement doit être disponible dans un format exploitable, afin de nous permettre de développer nos propres analyses comme il convient. Enfin, notre ambition concerne les finances sociales elles-mêmes, au travers de l'instauration d'une règle d'or. L'Assemblée nationale propose un compteur des écarts.

ce dispositif, déjà adopté l'année dernière, mes chers collègues, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la dette sociale et à l'autonomie. Il s'agit de prévoir que les comptes de la sécurité sociale affichent un équilibre sur cinq ans, afin de cesser de creuser éternellement la dette sociale que nous ambitionnons, depuis vingt-cinq ans, de ne pas transmettre à nos enfants. Bien sûr, un tel dispositif ne pourrait s'appliquer qu'à la sortie de la crise actuelle. Nous proposons donc que cette contrainte ne s'applique qu'à compter de la période 2024-2028, mais nous sommes naturellement ouverts à vos propositions,

Je conclus, madame la ministre, en répétant que nous abordons cette discussion dans un esprit constructif. Convenons-en, il serait très regrettable et contraire à tous les précédents en la matière qu'un texte portant sur un sujet aussi institutionnel, issu d'une proposition de loi de surcroît, ne fasse pas l'objet d'un vote consensuel entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour autant, un accord ne peut se faire à n'importe quel prix, et la seule avancée pour le Parlement de ces textes ne peut se résumer au droit de constater plus tôt dans l'année, dans une Lacss, que le Gouvernement s'est affranchi des objectifs fixés par le

ses yeux, « politique », par opposition à un texte technique ou anodin. Je lui en donne acte, mais, plus que d'un texte politique, je parlerai quant à moi d'un texte institutionnel. Il s'agit en effet de déterminer comment s'organisent les rapports entre les pouvoirs publics en matière de comptes sociaux. Il s'agit en particulier d'appliquer à ces comptes l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. En ces temps d'affaiblissement du consentement à l'impôt, voire de jacquerie fiscale moderne, mesurons l'importance du sujet, appliqué à 500 milliards d'euros de dépenses publiques Il s'agit donc concrètement de préciser la portée du vote que nous émettons chaque année dans cet hémicycle sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Historiquement, ce jeune texte, qui n'a que vingt-cinq ans, alors que le budget de l'État est la mère des parlements, est le fruit d'un compromis. Après l'accumulation des premiers déficits et le recours plus marqué à l'impôt pour financer la sécurité sociale, l'intervention des pouvoirs publics était bien sûr nécessaire, mais la prédominance d'un financement par cotisations, fondement de la gestion paritaire, ne semblait pas devoir laisser place à un véritable « budget » de la sécurité sociale. D'où les termes constitutionnels de « prévisions de recettes » et d'« objectifs de dépenses », censés ménager une place au caractère évaluatif de certaines dépenses. L'intention du constituant, puis du législateur organique, était pour autant très claire : la loi de financement de la sécurité sociale n'est ni une pétition de principe, ni une résolution, ni une loi de programmation. Elle a bien une portée normative, qui doit s'imposer à tous. Au fil du temps, cette portée normative est apparue de plus en plus prégnante. Des Ondam systématiquement dépassés, nous sommes passés aux Ondam respectés et aux actions correctrices, en recettes et en dépenses, pour combler le solde, le fameux « trou de la sécurité sociale », dont chacun mesure bien qu'il n'est pas technique. Médecins libéraux, entreprises du médicament, fédérations hospitalières et syndicats ne s'y trompent pas : le PLFSS fixe bien des enveloppes sans droit de tirage illimité sur les finances de la sécurité sociale. C'est pourquoi le compromis des origines exige une actualisation, tant il a paru encore plus crûment avec la crise sanitaire que, loin de laisser une marge à la gestion paritaire, cette construction laissait, de fait, les mains libres au Gouvernement. Au fil du temps, la sécurité sociale est devenue l'opérateur des politiques sociales de l'État, qui lui a transféré un certain nombre de charges qu'il assumait jusqu'alors. La part des cotisations sociales représente, en 2021, moins de la moitié des ressources Pour autant, l'exécutif peut accroître très sensiblement les dépenses, y compris de manière pérenne, sans repasser par l'autorisation parlementaire, puisque cela n'est pas juridiquement nécessaire. Quel souverain d'Ancien régime n'en aurait pas rêvé ? Au travers des « clauses » de révision, la commission des affaires sociales propose de mettre fin à cette anomalie. D'aucuns reprochent au texte de la commission d'intégrer au PLFSS l'assurance chômage, privant du même coup les partenaires sociaux du pilotage du régime.

Le Sénat s'était opposé à ces réformes, mais il nous semble aujourd'hui qu'elles ne sont pas réversibles : les partenaires sociaux peuvent-ils rétablir 2,4 % de prélèvements sur les salaires ? Peuvent-ils, sans apport extérieur, régler une dette de près de 70 milliards d'euros ? Nous ne le pensons pas et nous souhaitons que le Parlement ait son mot à dire de cette intégration, nous invitons le Sénat à considérer la réalité des mécanismes institutionnels qui sont à l'oeuvre et qui ont, sous couvert d'écarter le Parlement pour ménager les partenaires sociaux, ont conduit en réalité à écarter tout autant ceux-ci C'est donc bien une forme de reconquête démocratique que nous vous proposons, sans nous contenter de la seule loi d'approbation des comptes proposée par l'Assemblée nationale, qui nous conduirait simplement à constater, à l'été- Jean-Marie Vanlerenberghe l'a souligné -, que le Gouvernement n'a pas fait ce que nous avions décidé. Effectivement, ce n'est pas un texte technique ; il a bien l'ambition de nous permettre, dans cet hémicycle, de poser des actes politiques. La parole

la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont entraîné une dégradation significative et durable des comptes publics. Les dépenses ont augmenté très fortement en 2020, avec une hausse de 96,4 milliards d'euros. La dette publique

les conséquences financières à long terme pour les finances publiques nous ramènent au laborieux défi de la soutenabilité de la dette, en constante progression depuis cinquante

le régime d'assurance chômage, sans remettre en question le rôle des partenaires sociaux ni le paritarisme. En matière de lisibilité, les informations requises en annexe des lois rectificatives seront simplifiées, afin de faciliter le recours à ces outils outils budgétaires, qui seront désormais systématiquement déposés en cas de dépassement de plus de 1 % des crédits adoptés. En ce qui concerne la temporalité de l'examen des comptes sociaux, distinguer dans le temps l'examen des comptes du dernier exercice clos de celui des comptes de l'année en cours et à venir. Ainsi, un nouveau projet de loi de résultat sera examiné au printemps, sur le modèle des projets de loi de règlement, afin de valider les tableaux financiers relatifs au dernier exercice clos, ce qui correspond à l'actuelle première partie du PLFSS. Enfin, le pilotage pluriannuel des finances sociales sera facilité par deux innovations : l'ajout d'un article liminaire dans la présentant les prévisions budgétaires des administrations de sécurité sociale pour chaque année couverte et la création d'un compteur des écarts entre les prévisions de dépenses, de recettes et de soldes décrites dans le PLFSS

pour prendre connaissance du PLFSS et exercer son droit d'amendement. Par ailleurs, il sera immédiatement informé en cas de rupture des équilibres votés.

la règle d'or devrait permettre de garantir l'équilibre des comptes sociaux sur une période de cinq ans, une fois la crise de la covid passée. Dans la mesure où il s'agit d'un système souple, autorisant les dépassements en cas de circonstances exceptionnelles, nous y sommes favorables. Toutefois, nous devrons veiller à la cohérence des objectifs fixés dans l'Ondam avec la dynamique des dépenses du secteur hospitalier,

fois par le Gouvernement, le Parlement et la Cour des comptes afin d'améliorer les lois de financement de la sécurité sociale. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires y est favorable. Bravo

fiscalisation des ressources, vote des recettes et dépenses, équilibre financier de chacune des branches -renforce le paradigme financier de la protection sociale et les outils de la contrainte des dépenses. Ces deux propositions de loi, ainsi que les amendements adoptés, poursuivent cette logique d'ajustement des dépenses aux prévisions de recettes, enveloppe contrainte sur laquelle échouent toutes nos propositions pour en élargir l'assiette afin de répondre aux enjeux de la transition démographique et de mettre en place une politique de prévention et de promotion de la santé, d'égalité des territoires et d'accès universel à la protection sociale. À quand un projet de loi partant de l'analyse des besoins de la population et des territoires, induisant un objectif national de recettes Faute de renouer avec la finalité de la protection sociale, le rôle de la tarification à l'activité (T2A) dans la crise de l'hôpital public, des services d'urgence aux soins palliatifs, n'est jamais questionné à la veille d'étendre cette modalité de financement à l'hôpital psychiatrique, déjà sinistré. Nous regrettons que notre amendement visant à poser le principe selon lequel le financement d'un établissement de santé par la T2A ne doit pas représenter plus de la moitié de ses ressources afin de lui permettre d'assurer ses missions de service public ait été jugé irrecevable. Cela démontre, s'il en était que la T2A est bien un outil de limitation des dépenses et non d'efficience et d'efficacité des soins. La rénovation du cadre organique ne vise qu'à limiter les dépenses, en cohérence avec un autre cadre : celui du traité de Maastricht. L'Assemblée nationale avait rejeté un amendement visant à réintroduire les recettes dans le cadre d'analyse pour laisser la possibilité « de jouer sur le levier des ressources et diminuer les écarts entre les prévisions et le réel Aussi approuvons-nous l'amendement adopté en commission tendant à rappeler que l'équilibre comporte bien deux composantes et permet l'information sur les écarts en matière de recettes. Le compteur des écarts sort ainsi de son hémiplégie, ce qui permettra de suivre l'impact dynamique de l'augmentation constante des dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Par ailleurs, un écart traduit non pas forcément une dérive du réel, mais une prévision souvent déconnectée de la logique des besoins. Nous défendrons un amendement de suppression de la règle d'or visant à garantir l'équilibre financier parfait sur cinq ans des comptes de la sécurité sociale.

De plus, dans un contexte de crise sociale et sanitaire, d'accroissement des inégalités, de la pauvreté et de la précarité, cette règle d'or est particulièrement décalée. Le groupe écologiste est également opposé à l'extension du périmètre des lois de financement de la sécurité sociale à l'assurance chômage. À la fin de l'année 2018 déjà, la lettre de cadrage du Gouvernement imposant aux partenaires sociaux une économie de près de 4 milliards d'euros

De même, nous sommes défavorables à l'introduction d'une annexe sur les régimes de retraite complémentaire obligatoires, volonté constante du Gouvernement de s'inviter sur la gestion paritaire autonome. Il serait temps, en revanche, d'évaluer sérieusement l'effet des exonérations sociales sur l'emploi et la trajectoire de transition écologique, sans laquelle les effets nocifs de la dégradation de l'environnement sur notre santé ne cesseront de s'aggraver.

Le contexte dans lesquelles elles s'inscrivent est exceptionnel : la crise de la covid a en effet provoqué une forte dégradation du solde de la sécurité sociale, faisant ainsi plonger le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à 38 milliards d'euros en en 2020 et à 34 milliards d'euros en 2021. L'occasion nous est ainsi donnée de revoir le pilotage des finances sociales et de conforter du même coup les principes qui ont présidé, voilà vingt-cinq ans, à la création des lois de financement Plusieurs rapports, dont celui du Haut Conseil du financement de la protection sociale relatif à la modernisation des lois de financement de la sécurité sociale, de la Cour des comptes ou de la Commission pour l'avenir des finances publiques,

Nous le constatons chaque année un peu plus sur ces travées. Il nous est donc proposé, dans un souci de lisibilité, de modifier le calendrier et la procédure d'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale en anticipant d'une semaine leur dépôt devant le Parlement et, surtout, en transférant certaines annexes dans une nouvelle loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, à l'image de la loi de règlement du budget. Dans ce même esprit, les observations faites par les caisses et les organismes pourront nous être directement transmises. L'ambition de ces textes est également de tirer parti de la pratique parlementaire et d'offrir une meilleure adéquation entre le champ des lois de financement et celui de la protection sociale.

la raison qui a conduit l'Assemblée nationale à étendre le champ du PLFSS à la dette des établissements du service public hospitalier, considérant que ses effets sur l'équilibre général des comptes sociaux justifient sa place au sein du domaine facultatif des lois de financement de la sécurité sociale. Notre commission a souhaité supprimer ce dernier ajout, de la même manière qu'elle avait rejeté, lors du PLFSS pour 2021, la reprise d'une partie de la dette hospitalière par la caisse d'amortissement de

Nous proposerons également de préciser le contenu des annexes et de supprimer certains ajouts, qui, nous semble-t-il, les alourdiraient au risque d'en affecter la lisibilité. Au-delà de la technicité et de la froideur apparente de ce texte, il faut peut-être rappeler l'enjeu de cette réforme. Il s'agit bien sûr, nous l'avons dit, d'améliorer l'information du Parlement et la qualité des débats. Il s'agit aussi d'assurer la soutenabilité des dépenses sociales dans un contexte inédit. L'enjeu est de taille. d'autant plus que la sécurité sociale a consenti des efforts considérables afin de préserver nos concitoyens de la crise de la covid, pour financer la vaccination et les tests, traiter les personnes infectées et protéger les personnes les plus à risque. Il le sera tout autant quand il faudra panser les plaies, notamment les moins visibles. Je pense aux Assises de la santé mentale qui ont ouvert aujourd'hui. Il le sera encore dans les années et les décennies à venir, alors que la population française continue de vieillir et que le rôle des politiques sociales en faveur de l'autonomie devient central. Je terminerai en rappelant la défiance qui, chaque jour, se manifeste à l'égard de nos institutions et de nos politiques. Renforcer l'intervention et le contrôle du Parlement sur les lois de financement de la sécurité sociale n'est évidemment pas de nature à y mettre fin. Cela va pourtant dans le bon sens.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, de par leur technicité, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui ne rencontreront probablement pas un écho formidable dans la presse ni dans la population. Il nous faudra d'ailleurs une bonne dose de pédagogie pour en expliquer la teneur. Il faut dire que, pour nous-mêmes, parlementaires rodés à l'exercice, le cadre d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ne se caractérise ni par sa clarté ni par sa simplicité. Il nous est demandé, chaque automne, de nous prononcer sur un budget colossal, de plus de 500 milliards d'euros, qui touche à la vie quotidienne et intime des Français.

Il nous est proposé ici d'actualiser le cadre dans lequel députés et sénateurs votent le budget de la sécurité sociale, cadre qui n'avait pas évolué depuis 2005. On ne peut qu'être d'accord avec ces objectifs : simplifier, clarifier et rendre plus efficientes les lois de financement et ce après dix-huit mois de pandémie qui ont vu les dépenses de l'assurance maladie exploser et notre système de santé s'adapter dans des délais et des périmètres inédits, sans qu'aucun projet de loi de financement rectificative ne nous permette d'en débattre. Il serait tout de même faux de réduire les lois de financement de la sécurité sociale à leur simple aspect financier. Si leur champ d'application se limite aux dispositions financières, ils sont toujours l'occasion de débats sur notre modèle de protection sociale,

Nous soutenons donc toutes les mesures qui permettront de faciliter leur examen par les parlementaires, notamment l'anticipation d'une semaine du dépôt du PLFSS à l'automne, qui sera la bienvenue. D'autres mesures de lisibilité et de simplification devraient permettre de lever des difficultés fréquemment rencontrées par les parlementaires. au recours facilité aux lois de financement de la sécurité sociale rectificatives en cas de modification, en cours d'année, des équilibres votés précédemment. Je pense aussi à la création d'une loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Lacss) qui permettra, dès juin, de dédier un temps à l'examen des dépenses de la sécurité sociale de l'année précédente. Il est clair que cette partie de notre travail est aujourd'hui trop vite expédiée puisque nous sommes tout naturellement tournés vers le budget de l'année à venir. Je pense par ailleurs au renforcement du pilotage pluriannuel des finances sociales, qui offrira une meilleure visibilité sur l'état des dépenses,

simplifier notre travail. Ces textes proposent donc d'autres mesures bienvenues, que je vous proposerai de compléter par trois amendements visant à inclure les représentants des fédérations hospitalières dans la fixation de l'Ondam établissements de santé et à améliorer l'information relative aux dépenses et recettes du secteur du médicament. concerne l'intégration, dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale, de dispositions sur la dette des hôpitaux, nous maintenons notre position : en 2020, nous estimions que le transfert de la dette des hôpitaux à la Cades était injustifié. Le Gouvernement s'était engagé à reprendre une partie de cette dette au nom de l'État, car les hôpitaux appartiennent à l'État et non à l'assurance maladie. Nous soutenons donc la suppression, par la commission, de l'intégration des mesures relatives à la dette hospitalière dans les lois de financement de la sécurité sociale.

L'idée est intéressante et le débat mérite d'être posé. Le groupe du RDSE s'était d'ailleurs prononcé en faveur d'une règle d'or dans le projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l'autonomie en juillet 2020. Nous sommes pour la rationalisation des dépenses, pour ne pas laisser filer la dette et pour ne pas la transmettre aux générations futures.

En réalité, ce texte ne vise qu'une seule chose : imposer de nouvelles mesures d'austérité. Je constate avec colère que la droite sénatoriale et le Gouvernement poursuivent avec la même constance la réduction des dépenses sociales, la remise en cause de la gestion paritaire des caisses de sécurité sociale, le renforcement de l'étatisation de notre système social en rapprochant toujours plus le budget de la « sécu » de celui de l'État. La crise sanitaire et la prise en charge des dépenses des entreprises par la sécurité sociale, compensées par l'État, semblent donner des ailes aux militants de la mise sous tutelle de la sécurité sociale par Bercy, sous le prétexte de renforcer le droit de regard du Parlement. Depuis quarante ans, la gouvernance de la sécurité sociale a évolué vers un effacement des pouvoirs des syndicats dans l'administration des caisses, vers un renforcement du contrôle du Parlement et, depuis 2005, vers le verrouillage des dépenses avec la création de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie. Cette évolution progressive conduit à remettre en cause l'autonomie de la sécurité sociale et à renforcer la mainmise de l'État. La création de la contribution sociale généralisée (CSG) a entraîné une fiscalisation des recettes et une remise en cause de la cotisation sociale comme fondement du système de sécurité sociale. Ainsi, en 2021, 100 milliards d'euros de recettes proviennent de la CSG et la moitié des dépenses de la branche maladie est financée par l'impôt. À cela s'ajoutent les exonérations de cotisations sociales, décidées par les gouvernements, qui ont atteint 200 milliards d'euros au total entre 2011 et 2017. Enfin, la création d'une cinquième branche pour la perte d'autonomie, entièrement financée par l'impôt la CSG et la journée de solidarité, constitue une étape supplémentaire dans la transformation de notre système de sécurité sociale en un système de protection sociale. de la pandémie de covid-19, le déficit de la sécurité sociale, qui est de l'ordre de 35 milliards d'euros pour 2021, sert d'argument au renforcement du contrôle du Parlement. Il s'agit uniquement de fermer davantage le robinet des dépenses, pourtant vitales pour la protection de nos concitoyens. Alors que notre Alors que notre pays est toujours en état d'urgence sanitaire en raison des difficultés que rencontrent les hôpitaux pour soigner tous les malades, le Gouvernement, soutenu par la le Gouvernement, soutenu par la droite, veut reprendre les politiques d'austérité, celles-là mêmes qui ont entraîné la fermeture des hôpitaux de proximité, la suppression de 100 000 lits en vingt ans, la dégradation des conditions de travail des personnels, la pénurie de médecins du fait du et l'arrêt des investissements en raison de l'endettement de l'endettement des établissements. En votant ce texte, vous effacez d'une main l'ensemble des conclusions qui ont pu être tirées des erreurs commises avant la pandémie de covid-19. Ce ne sont pas les modifications de la droite sénatoriale en commission qui vont inverser la tendance, au contraire. La commission a réintégré l'assurance chômage et les régimes de retraite complémentaire dans le périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale, alors même que cette disposition avait été unanimement par les organisations patronales et syndicales. La commission a également instauré une règle d'or, qui contraint les comptes sociaux à l'équilibre sur cinq ans. Or si cette règle avait été appliquée l'an dernier, le Gouvernement n'aurait pas pu prendre en charge l'indemnisation chômage des salariés des entreprises fermées pendant la pandémie. Est-ce vraiment votre projet ? Allez voir les restaurateurs, les cafetiers et l'ensemble des commerçants qui ont pu bénéficier de la prise en charge par l'État de l'indemnisation chômage ! Tous vous diront, avec raison, qu'ils rejettent votre règle d'or, soyez-en assurés. d'or, soyez-en assurés. Nous refusons ce texte, qui constitue une étape supplémentaire vers une remise en cause de notre modèle de sécurité sociale. Nous vous opposons un projet alternatif, qui rétablit la cotisation sociale comme socle du système, qui réintègre une gestion paritaire des caisses de sécurité sociale par des administrateurs élus par les assurés sociaux. Nous proposons un financement de la sécurité sociale dépourvu d'exonérations, mais assuré par des cotisations patronales et salariales, ainsi que par des revenus financiers. Enfin, la suppression de l'Ondam comme carcan budgétaire doit permettre de renouer avec un financement qui parte des besoins de santé selon les territoires et non d'une enveloppe fermée.

Et si le Gouvernement avait voulu peindre un tableau plutôt impressionniste, la commission des affaires sociales s'est chargée de mettre les points sur les « i ».

Il nous faut des indicateurs plus proches du réel et, en ce qui concerne le PLFSS, des prévisions sur l'évolution de la qualité des soins, des rémunérations, des conditions de travail dans les établissements, du nombre de lits, des stocks tactiques et stratégiques de matériel médical ou encore sur les pénuries de médicaments

l'exposé des motifs de cette proposition de loi référendaire sur son article 3 : « Les décisions de fermeture de lits hospitaliers ne peuvent pas être contingentées en fonction d'une évaluation basée sur la performance du système de soin ni au prétexte qu'ils ne répondent pas à des critères de rentabilité économique,

besoins. Certes, ce texte ne contient pas de dispositions révolutionnaires venant heurter de plein fouet nos principes, mais il trace un peu plus un chemin vers la réduction des dépenses de notre système de protection sociale. On voit bien qu'au lieu d'assumer clairement cette trajectoire, ce texte quelque peu sibyllin modifie, à petites touches, les règles du jeu pour en faire un outil au service de la seule maîtrise budgétaire. Nous le regrettons. Sur le renforcement de la pluriannualité, par exemple, il s'agit de pointer systématiquement les écarts entre les prévisions de dépenses des lois de programmation et celles non seulement de la loi de financement de l'année, mais aussi des quatre années à venir, dans une vision strictement comptable. de loi est donc éminemment politique, et ce d'autant plus qu'elle traite aussi de la place des corps intermédiaires dans le processus de construction du budget de la sécurité sociale. L'élargissement du périmètre du PLFSS, voulu par notre commission des affaires sociales, par l'intégration des régimes de retraite Agirc-Arrco et de l'Unédic dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale, est une mesure à laquelle nous sommes opposés. L'étatisation de la sécurité sociale- quasi complète sans l'assurance maladie -qui est en marche tend à réduire le rôle et les prérogatives des partenaires sociaux et mène doucement vers la fin du paritarisme, pourtant indispensable pour l'équilibre et la concertation sociale. peut-on regretter de ne pas avoir, comme en Allemagne, des syndicats soi-disant responsables et, dans le même temps, leur tirer le tapis sous les pieds en les privant d'outils de gestion importants ? Quel rôle voulons-nous laisser aux organisations syndicales dans notre pays ?

débat précédent sur les finances publiques. Elles s'inscrivent dans la continuité idéologique des lois relatives à la dette sociale et à l'autonomie d'août 2020. Pour mémoire, le Gouvernement avait fait le choix de faire supporter la dette liée à l'épidémie Pourtant, cette dette relevait non pas d'un déficit structurel de la sécurité sociale, mais bien de décisions politiques. Il eut donc été tout à fait légitime que celle-ci soit reprise par le budget de l'État.

il semblerait, au travers de ce texte, que le monde d'après ne soit, hélas ! pas très social. La parole

vous vous en doutez, particulièrement sensible aux volets de ces textes relatifs aux pouvoirs de contrôle du Parlement, qui portent, je le rappelle, sur plus de 500 milliards d'euros de dépenses publiques.

En effet, reconnaissons que l'examen de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale est aujourd'hui bien trop tardif. Le fait de disposer à l'avenir d'un rendez-vous spécifique, à la fin du mois de juin ou au plus tard en juillet, permettra au Parlement d'examiner en temps utile les documents annexés aux futures lois d'approbation des comptes de la sécurité sociale, d'effectuer les auditions nécessaires et, au bout du compte, de se prononcer

Je pense à la mention expresse de l'évaluation des effets financiers de l'évolution des dispositions législatives encadrant des prestations sociales parmi les renseignements d'ordre financier et administratif que les commissions des affaires sociales sont en droit de demander et, surtout, d'obtenir d'obtenir aux termes de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale. Je pense aussi à l'obligation de répondre aux commissions des affaires sociales dans un format exploitable,

J'espère, madame la ministre, que ces apports subsisteront après la première lecture au Sénat et, au-delà, à l'issue de la navette. Enfin, j'aurai l'occasion de défendre un amendement tendant à supprimer l'introduction dans la loi organique du Printemps de l'évaluation

sécurité sociale. Je tenais, en tant que président de la Mecss, à souligner le caractère surprenant, pour ne pas dire peu élégant, de la démarche. Je me demande quelle serait la réaction des députés si nous introduisions dans le texte des procédures propres au Sénat

madame la ministre,

Certains se sont étonnés, voire émus- je l'ai entendu -que cette proposition de loi organique ne soit pas seulement un texte technique. Mais, mes chers collègues, qu'y a-t-il de plus politique que les rôles respectifs du Gouvernement et du Parlement dans la gestion de la moitié de nos dépenses publiques ? Nous nous situons en réalité au coeur de nos missions.

financement de la sécurité sociale a consacré le rôle du Parlement en la matière. Si la révision constitutionnelle de 1996 a créé les lois de financement de la sécurité sociale en les distinguant des lois de finances à l'article 34 de la Constitution, aucune ambiguïté sur l'intention du constituant. Certains veulent voir dans ce texte une vague constatation de dépenses presque extérieures au Parlement. C'est une erreur et c'est se méprendre sur la mission que nous confie la Constitution.

regarde aussi, madame la ministre, en disant cela : les lois de financement de la sécurité sociale offrent une extrême souplesse en matière de gestion des crédits publics. Nous le savons et le Gouvernement le revendique comme un avantage opérationnel. Mais ne confondons pas souplesse et laxité. Je le dis clairement ici : ce n'est pas parce que la sécurité sociale, et non l'État, verse des crédits à un opérateur que celui-ci doit disposer du jour au lendemain d'un guichet ouvert, sans contrôle du Parlement.

Madame la ministre, l'approche retenue par le Gouvernement sur les lois de financement de la sécurité sociale lors de l'année 2020 nous a surpris et marqués.

M. le ministre Dussopt nous l'a dit et répété : le Gouvernement n'a pas déposé de collectif social, car il estimait que la loi organique ne l'y contraignait pas. point que nous divergeons profondément. Certes, le droit ne l'y obligeait pas, mais la situation financière de la sécurité sociale rendait cet exercice politiquement et démocratiquement incontournable.

La première clause concerne le plafond d'emprunt de l'Acoss : nous ne nous satisfaisons pas d'une simple information lors de son relèvement. Nous souhaitons que les décrets soient pris après avis de la commission des affaires sociales.

Il lui impose seulement de recueillir l'avis du Parlement sur les dépenses qu'il entend faire au-delà des montants votés par celui-ci. Cela nous semble être le minimum. La troisième clause concerne plus particulièrement les périodes de crise et découle d'un amendement dont je suis l'auteure. Ainsi, en cas de rupture des équilibres financiers votés, à défaut d'un collectif social, le Gouvernement devra à tout le moins présenter au Parlement un rapport détaillant les raisons des dérapages financiers et actualisant les prévisions en matière de crédits votés. Surtout, car notre position est celle de parlementaires souhaitant assumer leurs responsabilités, les commissions des affaires sociales devront se prononcer sur les orientations proposées par le Gouvernement. Cette proposition de loi est donc un texte soucieux des droits du Parlement : devons-nous nous en excuser ?

Je crois en la sécurité sociale, à son rôle dans notre pays : elle est le ciment de la cohésion nationale et un instrument de solidarité. Je crois aussi à sa fonction d'amortisseur social en temps de crise économique. C'est justement parce que je crois en notre modèle social que je considère que son équilibre financier est le gage de sa soutenabilité.

mais, surtout, les moyens à la disposition du Parlement pour autoriser et suivre l'exécution des dépenses sociales. Pour ce qui est des dépenses d'assurance maladie, j'estime que le temps est venu de tirer les conséquences des évolutions de notre système d'assurance obligatoire. L'évolution L'évolution des recettes de cette branche- avec la fin des cotisations salariales pour la maladie et le poids majeur de la contribution sociale généralisée -, le changement profond de la logique assurantielle qui prévalait avec la protection universelle maladie (PUMa), ainsi que le financement des agences sanitaires par l'assurance maladie après la débudgétisation de Santé publique France, nous obligent à reconsidérer la construction de l'Ondam et le contrôle du Parlement sur celui-ci. Qu'on le regrette ou que l'on s'en félicite, ces réformes successives ont fait de la Caisse nationale de l'assurance maladie non plus une caisse gérée paritairement et dont la mission principale est le versement de prestations légales aux assurés, mais bien un opérateur de l'État pour la mise en oeuvre de sa politique de santé. de santé. La sécurité sociale d'aujourd'hui est-elle toujours celle qui a été pensée en 1945 ? Sauf à ne pas vouloir honnêtement le reconnaître, force est de constater que l'Ondam mélange aujourd'hui, sous un même régime budgétaire, des dépenses d'assurance sociale et des dépenses d'intervention. Cela peut constituer un atout, particulièrement pour le Gouvernement, en termes de facilité de gestion. Soit ! Mais ce confort tout relatif n'a pas été conçu par le législateur comme une dispense d'autorisation parlementaire de la dépense, sous prétexte que sa finalité est sanitaire. Soyons clairs : fallait-il acheter des masques et des respirateurs en urgence ? Évidemment oui ! Aurait-on pu demander au Parlement d'ouvrir une ligne de crédits ou, à tout le moins, le consulter plutôt que de procéder par arrêté ministériel ? Bien sûr Devait-on augmenter les soignants à l'issue de la crise sanitaire ? Oui ! Pouvait-on au préalable demander au Parlement d'approuver une dépense pérenne de plusieurs milliards d'euros ? Oui également, c'est son rôle constitutionnel. Surtout, comment admettre que, alors que le Gouvernement a annoncé en juin dernier un dépassement de l'Ondam de près de 10 milliards d'euros par rapport au montant voté en décembre, nous devions attendre cette année encore le mois d'octobre pour en discuter dans cette assemblée

Dans notre démocratie, ce n'est pas parce que la sécurité sociale paie que le Gouvernement doit décider seul ! Ce n'est pas le sens de l'histoire et, surtout, tel n'était pas l'intention du constituant de 1996 lorsqu'il a créé les lois de financement de la sécurité sociale. Madame la ministre, les rapports sur le devenir de l'Ondam et le pilotage des dépenses d'assurance maladie se succèdent et le parfait outil n'est certainement pas encore disponible. Mais où sont aujourd'hui vos propositions en la matière ? La commission des affaires sociales du Sénat, elle, a fait des propositions dans ce texte et j'y souscris pleinement.

Nous demandons de pouvoir mieux les suivre, d'évaluer les besoins supplémentaires et le montant des dotations d'intérêt général. Tout le monde reconnaît la fonction stratégique de certaines agences sanitaires : nous demandons à pouvoir suivre plus finement l'exécution de leurs dépenses. L'assurance maladie est un poste de dépenses majeur c'est surtout l'incarnation d'une politique publique essentielle, dont nous voulons débattre au Parlement. Tel est l'objet de ce texte. La parole Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en examinant ces propositions de loi, nous devons garder à l'esprit les enjeux des lois de financement de la sécurité sociale. Je rappelle que le budget des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse représente plus de 550 milliards d'euros. En outre, le contexte dans lequel nous examinons ces textes est singulier : jamais la sécurité sociale n'a connu une détérioration aussi brutale et rapide de ses comptes. Depuis 2017, les modifications des relations financières entre l'État et la sécurité sociale ont notamment été symbolisées par la non-compensation par l'État de certaines exonérations de cotisations ou baisses des prélèvements sociaux. Il en découle des pertes de recettes évaluées à environ 5 milliards d'euros pour 2019 par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. De ce fait, la sécurité sociale s'est trouvée, début 2020, en situation de fragilité et exposée de manière inédite à tout choc exogène. Nous connaissons la suite : la crise sanitaire est survenue et, avec elle, la très forte dégradation des comptes sociaux. La sécurité sociale fait partie intégrante de l'identité même de notre pays. Les Français y sont attachés. Laisser filer les déficits revient à la mettre en péril. L'État ne peut en faire une variable d'ajustement de sa gestion des finances publiques. J'en viens au fond des textes pour soutenir deux propositions adoptées par la commission des affaires sociales, sur l'initiative de son rapporteur Jean-Marie Vanlerenberghe, dont je salue le travail. En premier lieu, j'approuve la mise en place d'une règle d'or. L'idée d'éviter que, à l'issue de la crise actuelle, de nouvelles dettes se forment pour la sécurité sociale va tout à fait dans le bon sens. Le système proposé permettrait par exemple d'autoriser des déficits sur une année, mais imposerait de rattraper les pertes au cours des années suivantes. permettrait de garder une certaine souplesse en laissant la possibilité de reconnaître des « circonstances exceptionnelles » et de déroger à la règle. Il nous semble que le Gouvernement ne peut qu'accepter cette proposition puisque, lui-même, dans le projet de loi instituant un système universel de retraite, prévoyait une nouvelle gouvernance pour le pilotage financier du futur système. Avec la création d'une règle d'or, les comptes devraient nécessairement être à l'équilibre sur une période de cinq ans, quitte à prendre des mesures d'économie pour y parvenir.

et le Parlement pourrait voter des mesures ayant une incidence financière sur le régime d'assurance chômage. Certains parlent d'étatisation. S'il s'agit bien d'une recentralisation du pilotage financier du régime d'assurance chômage, force est de constater que le processus a déjà débuté depuis plusieurs années. Depuis 2018, en effet, le Gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage, qui sert en quelque sorte de base de travail pour la négociation. Comme nous l'avons vu en 2019, le Gouvernement peut refuser un accord interprofessionnel et fixer lui-même, par voie réglementaire, les règles inhérentes au système d'assurance chômage. Cette situation n'est pas pleinement satisfaisante. Le Gouvernement y tient une place prééminente et dispose d'une sorte de « pouvoir du dernier mot », qui écarte à la fois le travail des syndicats et du Parlement. Prévoir un vote de la représentation nationale dans le cadre des lois de financement de La même logique prévaut en matière de financement, avec le remplacement des contributions salariales d'assurance chômage par une fraction de CSG et la compensation des allègements généraux sur les contributions des employeurs.

Au-delà de ces mesures, nous partageons la volonté d'améliorer l'information et d'étendre les moyens de contrôle du Parlement. Le groupe Les Républicains apportera donc son soutien aux propositions de loi telles que la commission les a modifiées.